J’indique que M. le président du Sénat, Gérard Larcher, ne peut présider notre séance, car il est actuellement en Nouvelle Calédonie avec Mme la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun Pivet, pour une mission exploratoire de concertation et de dialogue. J’excuse également l’absence de M. le Premier ministre, qui effectue un déplacement à Bruxelles pour y rencontrer Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun d’entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. « Quand tu es à 38 jours de

sol. Désormais en première ligne, elle ne s’y est pas préparée et n’a aucune stratégie globale. Depuis des années, les Américains nous pressent de prendre une plus grande part du fardeau sécuritaire. Nous avons continué à croire que leur parapluie serait éternel nous sommes aujourd’hui seuls ou presque face à des ennemis qui menacent nos projets, nos valeurs et, surtout, notre sécurité. L’arrivée de 12 000 soldats nord coréens en Europe, après le soutien massif de la Chine et de l’Iran, marque un tournant dans la guerre. La réaction de la France ?

Si les États Unis et la Russie choisissent de négocier ensemble et par dessus notre tête le dépeçage de l’Ukraine et l’avenir de l’Europe, comment comptons nous réagir ? Si le retrait américain se confirme, avons nous prévu d’accroître notre soutien à l’Ukraine, et par quels moyens ? Soutenez vous l’engagement de Friedrich Merz, probable futur chancelier allemand, de permettre enfin à l’Ukraine de frapper les bases d’où partent les bombes qui détruisent le pays ? Enfin, quels sont les moyens et le calendrier pour refaire de l’Europe, après quarante ans de déni, la puissance militaire qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être ? Il n’y a rien de plus dangereux que de croire que nous ne sommes pas en guerre contre des dictateurs qui le sont contre nous et qui le disent. Pourtant, depuis février 2022, nous avons consacré à la défense de l’Ukraine 2 euros, l’équivalent d’un café, par mois et par Français.

président Malhuret, mille jours après le début de son opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine a lamentablement échoué à atteindre ses buts de guerre. Il a sacrifié des centaines de milliers de vies russes dans une guerre dont l’intensité n’a pas de précédent dans notre histoire récente. Il s’est rendu coupable de faits de déportation d’enfants ukrainiens, qui lui valent un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, devenant le premier dirigeant d’un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies à se trouver dans cette situation. Enfin, il a asphyxié son économie, qui est aujourd’hui au bord du gouffre, au point de l’amener à s’agenouiller devant la Corée du Nord pour tenter péniblement de chercher du renfort pour continuer à pilonner l’Ukraine. Mille jours après le début de cette injustifiable je crois Donald Trump trop avisé pour abandonner les Ukrainiens en rase campagne. Ce serait avaliser la plus grande annexion territoriale de notre histoire depuis soixante Ce serait consacrer la loi du plus fort et précipiter l’ordre international dans le chaos. Ce serait oublier qu’aucune paix juste et durable ne peut être conclue dans le dos des Ukrainiens et par dessus la tête des Européens. Parce que, mille jours après le début de la guerre, le soutien de la France et de l’Europe ne faiblira pas, quelles que soient les décisions de l’administration américaine. Dans quelques jours, les soldats ukrainiens formés et équipés sur notre territoire national gagneront le front. J’irai, avec Sébastien Lecornu et un certain nombre de parlementaires, leur rendre visite dès demain. Dans quelques semaines, les Ukrainiens recevront 50 milliards d’euros de la part des pays du G7, leurs alliés, financés par les revenus d’aubaine tirés des actifs russes gelés. Et dans quelques mois, ce seront les Mirage français qui voleront dans le ciel de l’Ukraine. C’est aux Ukrainiens qu’il appartient de décider des conditions et du moment d’ouvrir des négociations de paix, et c’est la responsabilité de leurs alliés de leur permettre d’entrer dans ces négociations en position de force.

l’onde de choc des restructurations chez Michelin et Auchan, qui menacent aujourd’hui directement 4 000 emplois, n’est vraisemblablement que le signe avant coureur d’une déferlante bien plus importante de défaillances d’entreprises. Vous aurez à faire la lumière sur les raisons et les responsabilités de ces plans sociaux. En attendant, on parle de 150 000 destructions d’emplois en France et d’un chômage grimpant à 8 % l’année prochaine, si rien n’est fait. Vos hypothèses de croissance, fondées exclusivement sur la consommation des ménages, seraient, dans ce cas, déjà caduques et, bien sûr, le budget pour 2025 s’en trouverait gravement compromis. Êtes vous prêt, monsieur le ministre, à considérer que notre économie a besoin d’être soutenue par l’investissement public, à la fois pour doper la réalisation des projets des collectivités locales et des territoires, mais aussi pour soutenir la recherche et l’innovation qui, seules – seules ! –, nous permettront demain de tirer notre épingle du jeu dans la compétition internationale En outre, l’Europe doit s’engager davantage. Quelle stratégie proposerez vous à nos partenaires européens pour mieux défendre et protéger nos entreprises, nos emplois et nos savoir faire ?

Monsieur le sénateur Daubet, je vous remercie de votre question et de la manière dont vous l’avez formulée, parce que vous avez résumé les défis qui sont devant nous, avec une situation difficile sur le front de l’emploi et de l’industrie et des difficultés que nous devons regarder en face. Ma responsabilité n’est pas de commenter, ma responsabilité n’est pas d’annoncer, mais elle est, en lien avec

en effet, passe par l’innovation et le développement de l’industrie verte sur notre territoire. Je suis donc heureux de vous confirmer aujourd’hui l’intention du Gouvernement, après l’invitation de nombreux parlementaires, issus notamment de ces travées, de soutenir la décarbonation de notre industrie, avec 1,5 milliard d’euros supplémentaires en faveur de l’ensemble des territoires.

conclus sur la question de l’Europe, que vous avez mentionnée : nous devons, collectivement, sortir de notre naïveté européenne. Le monde nous invite, avec la manière dont les évolutions politiques se font aux États Unis

C’est dans ce contexte que la COP29 sur les changements climatiques a débuté, pendant laquelle les puissances du monde doivent s’accorder sur le sujet de la finance climatique, là où elles ont échoué pour la biodiversité. COP se déroule sous la présidence d’un État pétrolier, une dictature où règnent la répression et la corruption et où parler d’environnement vous vaut la prison. De quoi discréditer la nécessaire coopération internationale.

Or, en Europe, nombreux sont ceux qui veulent la mort du Pacte vert. En France, la biodiversité est en constant déclin. Nous attendons un engagement fort, un an après la présentation de la planification écologique, votre budget semble acter un renoncement. Pourtant, le 5 septembre dernier, M. le Premier ministre faisait grand cas du concept de dette écologique lors de sa prise de fonctions. Dans ce contexte inquiétant, quels moyens comptez vous réellement mettre en œuvre pour relever le défi écologique, acculés que nous sommes devant l’effondrement de la biodiversité et l’urgence climatique ?

Nous le savons, le dérèglement climatique est devant nous : en France, nous en vivons les épisodes chaque semaine au travers d’aléas climatiques majeurs : inondations, canicules, sécheresses ou mégafeux. Nous le vivons aussi de manière plus insidieuse, avec la perte de rendement agricole, par exemple. Mais nous nous le vivons aussi à l’international, avec des évolutions géopolitiques qui ne sont pas nécessairement favorables. Nous agissons d’abord au niveau national. Je rappelle que la France est l’un des premiers pays à s’être doté d’une stratégie nationale biodiversité (SNB) en ligne avec les accords de Montréal

– Kanaky. Monsieur le ministre délégué chargé des transports, tous les ans, nous battons le record de l’année la plus chaude jamais observée. Réduire les émissions du secteur des transports devrait donc être votre priorité. comme d’autres avant lui, votre gouvernement s’entête à liquider Fret SNCF, pliant sans combattre devant la décision de la Commission européenne. Dans ces conditions, comment tiendrez vous votre engagement de doubler la part du fret ferroviaire d’ici à 2030 ? Depuis l’ouverture à la concurrence en 2006, Fret SNCF a été affaiblie par plusieurs plans de restructuration : 10 000 emplois ont été supprimés ces quinze dernières années. L’entreprise publique est maintenant menacée par un plan de discontinuité à la suite des 5 milliards d’euros de soutien financier de l’État français, condamné par l’Union européenne. Fret SNCF, démantelée en deux sociétés, devra ainsi abandonner 23 lignes de train dédiées et ne pourra pas candidater pendant dix ans sur des sillons extrêmement rentables. Elle se séparera de locomotives et d’actifs immobiliers et 500 postes seront supprimés. Rien d’étonnant, donc, à ce que des préavis de grève soient déposés. Pourquoi accepter de telles sanctions ? Ce plan de discontinuité est un non sens écologique et économique dans un pays qui souhaite se réindustrialiser. Vous cassez un outil qui représente près de 60 % des marchandises transportées par train en France, alors que la mise en concurrence a échoué partout en Europe. Monsieur le ministre délégué, aurez vous le courage de vos ambitions et défendrez vous notre opérateur public de fret contre le dogme de la concurrence libre et non faussée imposé par Bruxelles ?

le sujet. La première, c’est que le fret a bénéficié au cours des années passées de 5 milliards d’euros d’aides illégales au regard du droit européen. Et ce n’est malheureusement ni

pour le fret ferroviaire, avec une augmentation pour le wagon isolé à hauteur de 100 millions d’euros. Le Premier ministre a demandé, dans le cadre du budget pour 2025, d’accroître l’effort du Gouvernement à hauteur de 30 millions d’euros, et 4 milliards d’euros seront consacrés

réplique. le ministre, je doute de la robustesse de votre dispositif. D’autres solutions sont possibles. Appliquons un moratoire, comme le recommandait le rapport parlementaire d’Hubert Wulfranc. Entamons de nouvelles discussions avec Teresa Ribera, commissaire européenne récemment nommée. Travaillons avec les organisations syndicales et les partenaires qui proposent des projets alternatifs pour développer le rail. Ne prenez pas le risque, monsieur le ministre, de jeter des milliers de camions supplémentaires sur nos routes

est non seulement problématique pour nos agriculteurs, mais aussi en contradiction avec nos engagements environnementaux. Le rapport de Stefan Ambec a démontré en 2020 que ses coûts écologiques seront supérieurs à ses gains économiques, et Greenpeace n’a cessé de dénoncer le risque majeur que représente cet accord pour le climat et la biodiversité. En effet, il ne garantit pas que les importations européennes en provenance des pays du Mercosur ne seront pas liées à la déforestation. Pis, en favorisant les exportations sud américaines de bœuf ou de biocarburants, il contribuera à l’accélérer. Au delà de la problématique de la déforestation, l’accord est dépourvu de toute exigence contraignante quant aux modes de production. Or les normes environnementales sont autrement plus lâches dans les pays du Mercosur que dans l’Union européenne. Ce nivellement écologique par le bas se fait au détriment de la planète. Pour y remédier, la France a tenté d’y intégrer de la réciprocité, des normes et des clauses miroirs, sans succès. En l’état, le traité est donc contraire à l’accord de Paris et à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Madame la ministre, vous qui avez réaffirmé, lors de votre audition au Sénat, vouloir lutter contre tout dumping écologique, opposerez vous le veto français à la conclusion de cet accord ? ? Surtout, refuserez vous, au nom de l’environnement, une adoption séparée de son volet commercial par la Commission

le Président de la République l’a rappelée à maintes reprises, pour les raisons que vous avez citées, qui tiennent tout d’abord au fond de cet accord. Celui ci, aujourd’hui, ne réunit pas les garanties suffisantes pour que l’ambition environnementale soit au rendez vous, mais aussi pour protéger nos filières agricoles. Vous l’avez dit, l’accord de Paris doit être un élément essentiel de l’accord avec le Mercosur. En cas de violation du premier, le second doit pouvoir être suspendu. Il doit aussi comprendre des clauses de sauvegarde des mécanismes de sanction lorsque les obligations environnementales ne sont pas satisfaites. Il doit également respecter les règles en vigueur, celles que l’Union européenne impose à ses producteurs, notamment en matière de matière de déforestation. Garantir que nos partenaires commerciaux respectent en tout point les contraintes qui pèsent sur nos producteurs est une question de cohérence et de justice. Mais une autre raison explique que nous nous opposions à cet accord en l’état : nous tenons à ce que la Commission respecte le mandat qui lui a été confié par le Conseil, c’est à dire de conclure un accord d’association soumis à l’unanimité des États membres et à la ratification par les Parlements

où en est la promesse de plein emploi du président Macron ? Où en est la réindustrialisation de la France, dont les gouvernements successifs se félicitent depuis 2017 ? Que dites vous aux 1 254 salariés de Michelin en Maine et Loire et dans le Morbihan et aux 2 389 salariés d’Auchan dans les Hauts de France ? Leur dites vous, à eux aussi, que c’est simple, qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du travail ? ce mépris de classe s’ajoute une réalité aujourd’hui bien sombre : notre industrie va mal. Je pense aussi aux 1 700 emplois menacés chez Sanofi, dans l’Oise et le Calvados, ainsi qu’aux 228 salariés de Duralex, sauvés par leur reconversion en coopérative. Votre gouvernement poursuit la politique délétère déjà en place depuis plusieurs années, avec 80 milliards d’euros d’allégements concédés pour les gros salaires et les grandes entreprises qui vont grever le budget de la sécurité sociale. Flexibilité de l’emploi, facilitation des licenciements : cela protège t il l’emploi ? Non. ? Non. Cela protège t il l’industrie ? Non. Pis, les gouvernements successifs ont, depuis 2017, dégradé les droits sociaux et pénalisé les chômeurs. Pour beaucoup, c’est la double peine. Il ne s’agit pas seulement de milliards d’euros, mais d’êtres humains qui peuplent notre pays et qui souffrent aujourd’hui autant qu’ils s’inquiètent de leur avenir et de leur famille. Étant née en Lorraine,… je sais ce qu’est le regard d’un enfant qui ne verra plus ses parents travailler. Victor Hugo disait : « Aidons, protégeons, secourons, avouons la faute publique et réparons la. » Il disait encore : « C’est du droit de tous les faibles que se compose le devoir de tous les forts. Madame la ministre, comment le Gouvernement compte t il enfin réparer sa politique pour protéger l’emploi industriel et anticiper les mutations à venir, notamment la mutation écologique et la décarbonation de l’industrie, dont la France ne peut se passer ? Merci…

en perspective et de rappeler ce qui a pu marcher dans notre pays. Mais vous avez raison, madame la sénatrice, les conditions économiques se durcissent, avec une accélération de la hausse du nombre de procédures collectives d’entreprises en difficulté.

et américaines. Toutes les réponses, je dis bien toutes les réponses, qu’elles viennent des ministères chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie comme du travail, doivent être mobilisées, que ce soit sur le plan

a consacré un chapitre assez important à l’épineuse question de la corruption. Les choses n’ont pas été faciles, car nous avons constaté que les administrations centrales et les inspections générales avaient peu de documents solides sur ce sujet, laissant entendre que le Gouvernement regardait cela d’un peu loin.

des informations sont recueillies et sont ensuite communiquées à des narcotrafiquants, moyennant rémunération. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous avez à plusieurs reprises utilisé le terme de « narco État ».

ministre de la justice. Le 14 mai dernier, à Incarville, dans le département dont je suis élue, l’Eure, l’attaque d’un fourgon pénitentiaire a fait deux morts et trois blessés. Elle a suscité une très vive émotion parmi les agents pénitentiaires et toute la population française. Six mois après, les agents pénitentiaires restent inquiets. Je salue leur courage, car ils œuvrent chaque jour pour la population carcérale. Je me suis rendue récemment à la maison d’arrêt d’Évreux, où était incarcéré Mohamed Amra. Elle affiche à ce jour un taux de surpopulation carcérale de 189 %, avec quatre détenus par cellule de 10 mètres carrés. ai constaté les conditions de travail difficiles des agents, qui exercent dans des locaux étroits et vétustes, malgré un plan de travaux pluriannuel. Cette maison d’arrêt a 112 ans

Leur constat est implacable : ils se considèrent comme les grands oubliés de l’administration. Il est urgent de replacer les personnels au centre de la prise en charge. La qualité de vie au travail des agents ne pourra s’améliorer que lorsque les conditions de détention auront évolué. Après le drame d’Incarville, un protocole d’accord pour renforcer la sécurité des agents a été signé par votre prédécesseur avec l’intersyndicale de l’administration pénitentiaire. Toutefois, les agents s’interrogent sur son application effective. des sceaux ? Il aura fallu le drame d’Incarville pour réfléchir à des mesures de sécurité réclamées depuis de nombreuses années par les agents. Vous avez récemment annoncé que l’objectif de construction de 15 000 places nettes de prison d’ici à 2027 ne sera pas atteint

et au centre de détention de Val de Reuil, sur l’état des prisons et les conditions de travail et de sécurité des agents de la direction de l’administration pénitentiaire Vous évoquez en particulier les suites données au protocole dit d’Incarville, après le drame que nous avons vécu : l’attaque d’un fourgon qui, vous l’avez rappelé, a entraîné la mort de deux personnes et fait trois blessés. Je tiens, comme vous, à saluer l’engagement sans faille des personnels de l’administration pénitentiaire. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et méritent tout notre soutien et notre solidarité – je ne les oublie pas.

Cela me permettra de respecter les engagements qui ont été pris vis à vis de ces personnels. Les 33 mesures contenues dans ce protocole sont en cours de mise en œuvre

que les leçons des crimes de la France dans ses prétendus territoires d’outre mer ne seraient pas complètes sans mentionner les récentes violations des droits de l’homme par le régime. Rappelons que l’agitation a été entretenue en Nouvelle Calédonie et en Afrique par le Groupe d’initiative de Bakou

du conflit du Haut Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Pensons à ces plus de 100 000 personnes déplacées qui ont dû fuir leurs terres ancestrales. Madame la ministre, à l’heure où l’Europe et la France sont bafouées, je pense qu’il faut avoir le courage de faire la politique de la chaise vide.

à Bakou sont inacceptables. Scandaleux, oui ! Les attaques directes contre notre pays, ses institutions et ses territoires sont injustifiables. L’Azerbaïdjan instrumentalise la lutte contre le dérèglement climatique pour suivre un agenda personnel

Les propos tenus par les autorités de ce pays en faveur des énergies fossiles sont également inacceptables, alors que les diplomaties française et européenne avait obtenu un accord universel sur la sortie progressive des énergies fossiles de la COP28. Cela est indigne d’une présidence de COP. À l’inverse, je veux saluer le Brésil et le Royaume Uni, qui ont pris l’engagement de revoir à la hausse leur trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre. C’est de cette dynamique positive, et non d’une attaque d’une déplorable bassesse, que la communauté internationale a besoin pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Compte tenu de cette situation nouvelle,

que les équipes de négociations françaises ne ménageront pas leurs efforts, avec mon appui à distance et en lien avec nos partenaires européens, pour protéger la planète et nos populations. Nous continuerons à plaider pour le plus haut niveau d’ambition dans la mise en œuvre de l’accord de Paris, dont nous sommes les gardiens, dix ans après son obtention.

trouveront encore en première ligne, demain, pour redresser notre pays face à la crise économique et budgétaire qui va s’abattre sur nous. Ils méritent mieux que les clichés éculés, alors que le ministre de la fonction publique, dans une forme de trumpisme à la française, n’a rien trouvé de plus judicieux que de s’acoquiner avec Elon Musk,

La parole est à Mme Jacqueline Eustache Brinio, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le ministre, vous avez tenu à saluer le courage de cette jeune femme, qui a commis là un acte de résistance et s’est hissée au rang d’icône. Avez vous des informations sur ce qui est advenu d’elle et avez vous eu des contacts avec l’ambassade d’Iran ?

vous l’avez rappelé, des ténèbres obscurantistes dans lesquelles l’Iran est aujourd’hui plongé a surgi une icône du combat des femmes iraniennes. Ce combat, c’est celui de Mahsa Amini, des centaines de femmes tuées dans la répression sanglante des manifestations par le régime, des milliers de femmes emprisonnées ou vivant dans la peur de la répression. C’est bien sûr celui du mouvement « Femmes, vie, liberté », de toutes les femmes iraniennes qui aspirent légitimement à la liberté et à la dignité.

Une icône pour toutes celles et tous ceux qui résistent à l’obscurantisme, parfois au péril de leur vie, qui défendent inlassablement les droits de l’homme, des femmes, et des enfants.

que s’amplifier. Le régime des mollahs et le corps des gardiens de la révolution islamique ont exécuté, très majoritairement par pendaison, plus de 800 personnes en 2023,

pour traiter le problème du dévoilement chez les femmes, nos craintes sont légitimes concernant Ahou Daryaei. Rendons hommage au courage de toutes ces femmes – Mahsa, Ahou et tant d’autres – qui se battent pour faire valoir leurs droits, sous un régime islamique qui veut les invisibiliser. Trop de femmes sont victimes d’un véritable apartheid sexuel

Ma question s’adresse à M. le ministre délégué chargé des transports. Si le Gouvernement doit faire face actuellement à des appels à la grève, il en est un qui a un air malheureusement trop connu, celui du traditionnel chantage à la grève de Noël à la SNCF.

On pourrait débattre à l’envi des défis ferroviaires, mais, en définitive, les usagers du mois de décembre n’y seront pour rien : ils souhaiteront simplement retrouver leur famille à la veille de Noël.

Oui, le droit de grève est un droit constitutionnel ; c’est pourquoi nous n’acceptons pas de le voir détourné, et encore moins dévoyé.

pour les usagers de la SNCF. La continuité du service public est un principe constitutionnel au même titre que le droit de grève. Je suis également attaché à chacun de ces deux principes.

dépit de la prise de conscience du rôle central joué par les départements, ces derniers subissent une asphyxie budgétaire insoutenable. Selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2023, les départements sont l’échelon de collectivité territoriale

et dépourvus d’un levier fiscal pour accroître leurs recettes, les départements, acteurs clés de la justice sociale et de la résilience territoriale, voient leur rôle gravement compromis.

je connais votre détermination, monsieur le ministre, il reste que chacun doit agir dans le même sens. Il nous faut transcender les clivages et combattre les discours portés par une idéologie qui nie les violences, voit dans l’insécurité un simple sentiment et s’offusque dès que le mot « répression » Dans la ville natale de Victor Hugo, ces démagogies dépassent l’imaginable, car même si les polices municipales, en appui, ne sont pas la solution à tous les problèmes, elles doivent jouer leur rôle et être utilisées dans toute l’étendue de leurs compétences. Peut être faudrait il s’assurer qu’un maire ne puisse pas vider sa police municipale de toute efficacité en la privant d’armement. La priorité que nous devons donner à nos concitoyens est à ce prix et parfaitement conciliable avec la libre administration des collectivités locales. Il nous faut également développer partout la vidéosurveillance, encore trop souvent refusée alors qu’elle est un appui inestimable dans le travail de la police et de la justice. Ma question est simple, monsieur le ministre pouvons nous durablement accepter qu’un maire interdise à sa commune et à sa population les moyens de l’efficacité pour leur sécurité ?

Le 8 octobre, elle a ouvert une nouvelle procédure devant l’OMC, concernant cette fois les droits provisoires appliqués par la Chine sur les brandies, et donc sur le cognac. et donc sur le cognac. La ministre Sophie Primas, bien connue au Sénat, s’est rendue du 3 au 6 novembre dernier à Shanghai pour rappeler avec fermeté aux autorités chinoises notre détermination à défendre nos filières contre ces droits de douane illégitimes.

Trois ans plus tard, les habitants et les élus attendent la concrétisation totale de cette promesse présidentielle qui engage autant Emmanuel Macron que ceux qui ont contribué à le faire réélire. donc aujourd’hui ? Selon le projet de loi de finances pour 2025, les quelques crédits inscrits pour le renouveau du bassin minier participeraient à clôturer les financements précédents, sans nouvel engagement financier de l’État.

minières ? Les collectivités ont besoin d’être rassurées sur la participation financière de l’État à leurs projets de réhabilitation. Notre territoire fut jadis considéré comme possédant le plus beau logement social du monde.

en moyenne, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents ; il a été observé une augmentation de 16 % des violences intrafamiliales non conjugales entre 2020 C’est peu dire que ces chiffres vertigineux et glaçants nous imposent une démarche volontariste et active en faveur de la défense et de la protection de notre jeunesse. Les impacts de ces violences sur les enfants sont nombreux ; je pense à leur santé mentale et physique, leur vie affective, à leur scolarité, mais aussi, plus largement, à leurs relations sociales. Les professionnels de la protection de l’enfance alertent depuis de nombreuses années sur l’urgence des situations et l’insuffisance des actions de nos institutions, qu’il s’agisse des réponses judiciaires, des moyens budgétaires ou encore de l’arsenal législatif.

Bien entendu, en grandissant, il leur arrive de témoigner. Tout le monde se souvient, par exemple, de la parution du livre de Camille Kouchner, mais ces témoignages restent rares et arrivent souvent trop tard. Le cas de l’inceste est peut être le symptôme le plus évident des carences de notre système, puisque, encore aujourd’hui, il demeure très faiblement condamné, soit pour des motifs de prescription, soit faute de preuve. Un tel constat est inadmissible, d’autant qu’il place les victimes dans une forme de précarité juridique qui profite aux agresseurs. L’évolution récente des lois pénales et civiles relatives aux violences faites aux enfants témoigne d’une prise de conscience de notre société. Européen avait déjà souhaité alerter les pouvoirs publics sur les carences de notre législation, en déposant le 30 septembre 2019, sur l’initiative de notre ancienne collègue Françoise Laborde, une proposition de résolution visant à engager diverses mesures pour intensifier la lutte et la prévention contre l’inceste et à demander sa surqualification pénale. Deux années plus tard, sur l’initiative d’Annick Billon, le Sénat s’était engagé dans cette voie.

plus encore lorsqu’ils sont incestueux. Dans la continuité de ces travaux, la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a entretenu cette dynamique, en instituant de nombreux dispositifs attendus

permettant au juge aux affaires familiales (JAF) de statuer en urgence, entre autres mesures, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste parental vraisemblable. Seulement, je souhaiterais aller au delà de cette préconisation, en couvrant tout fait de violence susceptible de mettre en danger l’enfant et non pas seulement les violences incestueuses. Bien entendu, nous savons qu’il existe déjà de nombreux moyens qui permettent aux pouvoirs publics d’agir en cas de maltraitance. Le juge des enfants peut, par exemple, émettre des ordonnances de placement. Il existe également l’assignation à bref délai, qui permet au juge aux affaires familiales de se prononcer dans l’urgence, sous quinze jours, notamment en cas de violences à l’égard de l’enfant. Enfin, citons l’ordonnance de protection et l’ordonnance de protection provisoire, dont les mesures peuvent également bénéficier aux enfants. Nous comprenons donc que l’ajout d’un nouveau dispositif puisse poser certaines difficultés, mais il faut reconnaître que l’architecture actuelle souffre d’une forme de dispersion et qu’il n’existe pas de moyen unique spécifiquement consacré à la protection des enfants dans l’urgence, comme c’est le cas actuellement en matière de violences conjugales. Aussi, nous avons considéré qu’il était pertinent d’envisager la création d’un nouvel outil, qui, d’une certaine manière, regrouperait tous les autres. Cela permettrait de mieux prendre en compte la spécificité de ces violences,

m’a indiqué – elle vous le précisera sûrement d’ici quelques instants – que, dans leur grande majorité, les acteurs de la protection de l’enfance n’étaient pas nécessairement favorables à la création d’un nouvel outil.

Seulement, le dispositif inspiré de l’ordonnance de protection qu’elle tend à insérer dans le cadre juridique actuel suscite une grande réserve, quasi unanime, chez les acteurs de la protection de l’enfance que j’ai entendus Les magistrats concernés, qu’il s’agisse des juges des enfants, des juges aux affaires familiales ou des procureurs de la République, mais aussi les avocats, les services de la Chancellerie, une partie des associations consacrées à la protection de l’enfance et même, dans une certaine mesure, la Ciivise, pourtant à l’origine de la proposition, soit y sont opposés, soit conditionnent leur soutien à des modifications tellement substantielles qu’elles dénatureraient le dispositif du texte. Cela tient à deux raisons principales principales : les défauts juridiques de cette ordonnance de sûreté ; le fait qu’elle altérerait la lisibilité et l’efficacité de la protection judiciaire de l’enfance. En conséquence, il ressort des travaux de la commission des lois qu’un tel dispositif nuirait à l’objectif que l’auteure de ce

outre moins favorables que celles des autres dispositifs de protection de l’enfance, qui seront brièvement exposés par la suite. Par ailleurs, cette saisine n’exigerait pas le dépôt d’une plainte pénale, ce qui est contraire au devoir de protection qu’un parent doit à son enfant. le dispositif ne prévoit pas de sanction en cas de méconnaissance de l’ordonnance, ce qui la priverait d’effectivité. En outre, il serait permis au juge de retirer tout ou partie de l’autorité parentale et non d’en suspendre seulement l’exercice cette mesure, d’une particulière gravité, paraît tout à fait inadaptée à une procédure d’urgence qui ne conclut pas à une reconnaissance de culpabilité. Enfin, ce dispositif étendrait indûment l’office du JAF, auquel il n’incombe pas, en principe, de se prononcer sur une potentielle infraction C’est ce que je souhaite aborder en second La protection judiciaire de l’enfance repose sur plusieurs procédures, qui sont adaptées à la situation de l’enfant présumé victime de violences. Nous pouvons, pour simplifier, répartir les dispositifs en deux catégories principales : d’une part, ceux qui permettent d’assurer la protection judiciaire d’un enfant en l’absence d’un parent protecteur et, d’autre part, celles qui fournissent à un parent protecteur les moyens de protéger son ou ses enfants. En l’absence d’un parent protecteur, la protection judiciaire de l’enfant présumé victime de violences repose en principe sur l’action du juge des enfants. Ce dernier peut, en effet, prendre des mesures dites d’assistance éducative, parmi lesquelles figurent notamment l’ordonnance de placement ou, exceptionnellement, la détermination des droits de visite et d’hébergement des parents. Notons que ces mesures peuvent être ordonnées en urgence par le procureur de la République, dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire. Le procureur doit ensuite saisir, sous huit jours, le juge des enfants au delà des mesures qu’elle permet d’obtenir, la saisine du juge des enfants est protectrice en elle même, grâce aux diverses garanties procédurales qui l’accompagnent et qui témoignent de la spécialisation de ce juge. Un parent protecteur peut, par ailleurs, recourir à plusieurs dispositifs qui assurent la protection judiciaire d’un enfant présumé victime de violences. Considérons, en premier lieu, la saisine générale du JAF, ouverte à l’un des parents ou au ministère public, afin qu’il se prononce quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. À cette saisine générale s’adjoint une procédure d’urgence mise en œuvre sous quinze jours, l’assignation à bref délai, qui figure à l’article 1137 du code de procédure civile. Le code civil prévoit par ailleurs la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement d’un parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par un juge d’instruction. La loi du 18 mars 2024 a d’ailleurs récemment étendu les motifs de cette suspension.

Seulement, j’ai voulu poursuivre mes échanges avec les acteurs de la protection de l’enfance et l’auteure de la proposition de loi, notre collègue Maryse Carrère, afin de dégager une solution favorable à la protection de l’enfance. Je le répète, seul l’objectif consistant

Ils visent, en un mot, à étendre le dispositif existant de l’ordonnance de protection aux cas dans lesquels seul l’enfant est présumé victime de violences. Nous aurons bien entendu l’occasion d’y revenir lors de leur examen, mais permettez moi d’observer d’ores et déjà qu’ils apportent une réponse à l’essentiel des problèmes juridiques que soulèverait l’ordonnance de sûreté : les conditions de saisine seraient harmonisées ; un dépôt de plainte pénale serait requis lorsque les violences concernent un enfant ; le dispositif prévoirait une sanction ; seul l’exercice de l’autorité parentale pourrait être suspendu ; l’office du JAF serait mieux respecté. ces amendements permettrait donc de limiter les risques que posait initialement la proposition de loi quant à la lisibilité du cadre juridique actuel de la protection de l’enfance et du fait des défauts juridiques précités.

Deux choses nous paraissent certaines : la première, je le répète, c’est notre attachement partagé à la protection des enfants ; la seconde, ce sont les qualités du travail parlementaire, l’exemple de cette proposition de loi l’atteste. Nous avons pu, grâce à nos échanges, éclairés par des auditions et consultations ouvertes, auxquelles de nombreux sénateurs de divers groupes ont participé – qu’ils en soient remerciés –, souligner les défauts d’un dispositif et en imaginer un autre. Ce dernier connaît cependant encore des limites. Le travail parlementaire, notamment lors de l’éventuel examen du texte à l’Assemblée nationale, permettra de les identifier et de les corriger. Madame la ministre, je ne doute pas de votre attention. Nous le savons tous ici, la cause des mineurs doit être traitée comme une cause majeure ; les enfants resteront notre priorité, inlassablement. La parole

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, madame l’auteure de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd’hui un texte visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. auteure souhaite créer, sur le modèle de l’ordonnance de protection prévue à l’article 515 9 du code civil, un dispositif spécifique de protection des enfants victimes de violences ou de violences sexuelles incestueuses : l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Ce dispositif s’ajouterait à ceux qui existent déjà en droit positif, tout en présentant des spécificités. Ainsi, selon ce nouveau régime, inscrit dans un titre dédié du code civil, l’ordonnance de sûreté pourrait être délivrée dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fixation de la date de l’audience, « lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence susceptibles de le mettre en danger, commis par une personne titulaire sur celui ci d’une autorité de droit ou de fait, et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise La délivrance d’une ordonnance de sûreté permettrait le prononcé, pour une durée de six mois, de mesures provisoires restrictives de liberté, telles que des interdictions de contact et de et de paraître, le port d’un dispositif électronique mobile antirapprochement permettant la géolocalisation permanente du parent violent et de son enfant, ou encore le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de l’exercice L’objectif de cette proposition de loi est particulièrement louable, puisqu’il vise à améliorer la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. Cette protection, vous le savez, est une priorité absolue pour le Gouvernement. Je rappelle à ce titre que, le 20 novembre 2023, un plan de lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2023 2027 a été lancé, qui s’articule autour de vingt deux actions tendant à améliorer la prévention des violences et la protection des enfants.

Cette loi, directement inspirée des recommandations de la Ciivise, permet aux magistrats de remettre en cause plus facilement les droits parentaux du parent poursuivi ou condamné pour des faits de viol ou d’agression sexuelle incestueux commis sur son enfant. Elle permet ainsi la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement dès le stade des poursuites ; elle crée un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de viol ou d’agression sexuelle incestueux elle prévoit le retrait obligatoire de la titularité de l’autorité parentale en cas de condamnation pour viol ou agression sexuelle incestueux. garantit une protection efficace à l’enfant victime, en empêchant le parent agresseur de continuer à entretenir des liens avec lui et de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de celui ci. Il rappelle, en creux – puisque le dispositif se greffe sur la procédure pénale –, que, en cas de faits délictuels ou criminels commis par un parent à l’égard de son enfant, nos règles de procédure pénale intègrent une dimension de protection de l’enfant. Ainsi, si les éléments de l’enquête confirment, à l’issue de la garde à vue, l’existence d’indices graves et concordants ou la caractérisation des faits commis, le parent mis en cause peut être placé sous contrôle judiciaire, voire en détention provisoire, permettant son éloignement et la protection de l’enfant. c’est la procédure pénale qui doit, en première intention, permettre d’assurer la protection de l’enfant victime. Il me paraît fondamental de le rappeler, au regard de la gravité des faits, pour lesquels le dispositif soumis à la discussion aujourd’hui est prévu. que je comprenne et partage bien entendu la volonté de toujours mieux protéger nos enfants, il ne me semble pas que cette proposition de loi puisse contribuer Le dispositif qu’elle crée, sur lequel je me dois d’émettre d’importantes réserves, est en effet moins efficace que le droit existant. Je m’explique. Lorsque l’enfant est victime de violences physiques ou sexuelles de la part de l’un de ses parents, indépendamment de la procédure pénale qui devrait être engagée sans délai au regard de la nature des faits, tant le juge aux affaires familiales que le ministère public chargé des mineurs et le juge des enfants, spécialisés dans la protection des enfants en danger, peuvent d’ores et déjà intervenir en urgence, et parfois même sans délai. à l’autre parent, qui est le premier protecteur de l’enfant en tant que titulaire de l’autorité parentale, il peut déjà saisir le juge aux affaires familiales en urgence, dans le cadre de la procédure de l’assignation à bref délai, qui permet d’obtenir une date d’audience rapidement, et même en extrême urgence dans le cadre de la procédure de référé, qui permet, elle, d’assigner à heure indiquée, y compris les jours fériés ou chômés. Ces procédures permettent au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur, exactement comme il est proposé de le faire au travers de cette ordonnance de sûreté, et ce dans un délai beaucoup plus rapide, avec le référé d’heure à heure. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les violences commises sur l’enfant s’inscriraient dans un contexte de violences intrafamiliales avec des violences au sein du couple, l’ordonnance de protection délivrée au parent victime de violences profite également à l’enfant. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales peut prononcer des interdictions de contact entre le parent et l’enfant, et peut statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et le sort du logement familial. De leur côté, le procureur de la République ou le juge des enfants ont déjà la possibilité de prendre, sans délai et à toute heure du jour et de la nuit, au besoin avec le concours de la force publique, une ordonnance de placement provisoire qui permet d’extraire immédiatement l’enfant de son domicile sans débat préalable. Le cas échéant, l’enfant peut être placé chez l’autre parent et les droits de visite et d’hébergement du parent agresseur peuvent être réservés. L’enfant est ainsi immédiatement protégé. Vous l’aurez compris, en permettant au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur l’exercice de l’autorité parentale et le sort du logement familial, et au procureur de la République ou au juge des enfants d’extraire immédiatement l’enfant de son milieu familial, notre droit dispose déjà d’un arsenal juridique efficace pour protéger en urgence l’enfant victime de violences intrafamiliales. Ainsi, confier au juge aux affaires familiales une compétence concurrente à celle du juge des enfants, qui est le juge naturel en matière de protection de l’enfance, conduirait à une perte de lisibilité de notre organisation judiciaire. Ce sont ces éléments de réflexion que nous devrons avoir à l’esprit lorsque nous examinerons les amendements, dont celui de Mme Carrère, qui ont en remplacement du dispositif de l’ordonnance de sûreté, le dispositif de l’ordonnance de protection, lorsqu’il paraît vraisemblable que l’enfant a subi un viol ou une agression sexuelle incestueux ou des faits de violence de la part de l’un de ses parents ou de l’un de ses beaux parents, en cas de cohabitation. Je comprends que ces amendements visent à corriger certaines difficultés rédactionnelles et procédurales du texte initial et c’est positif, car notre droit, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les victimes les plus vulnérables, doit être clair et efficace. L’enjeu est trop important. Les critères sur lesquels reposerait le prononcé d’une ordonnance de sûreté manquent d’objectivité, qu’il s’agisse de la condition selon laquelle « il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise » ou de celle selon ou de celle selon laquelle la commission des faits jugée vraisemblable doit être « susceptible » de mettre l’enfant en danger. Par ailleurs, concerne le dispositif électronique mobile antirapprochement, qui est l’une des mesures de l’ordonnance de sûreté proposée initialement, la rédaction nécessite des éclaircissements, car elle laisse entendre que tous les mineurs pourraient en bénéficier, alors même que ce dispositif nécessite d’en comprendre pleinement le fonctionnement et que sa généralisation pourrait mettre les enfants en situation de conflit de loyauté. Enfin, le texte cite, parmi les effets de l’ordonnance de sûreté, la possibilité pour le juge aux affaires familiales de retirer la titularité, et non le simple exercice, de l’autorité parentale. Je rappelle que cette prérogative est en principe confiée non pas à un juge seul, statuant dans l’urgence, mais à un tribunal composé de trois juges, en raison de la gravité de cette décision. Tous ces arguments m’amènent à exprimer des réserves importantes sur ce texte, malgré, encore une fois, le but plus que louable qu’il vise et auquel je m’associe.

à celles qui existent déjà, c’est à la lisibilité du droit et à l’accès au juge que l’on porterait atteinte. Conservons une vision d’ensemble sur les outils existants de protection des mineurs. N’ajoutons pas de la complexité à des situations déjà terriblement compliquées. Gardons de la cohérence pour que la protection soit

mes chers collègues, nous pouvons tous en convenir, malgré de nombreux progrès accomplis au cours des dernières années au sujet des violences intrafamiliales, les violences commises spécifiquement sur les enfants sont encore bien trop nombreuses. La Ciivise avance ainsi le chiffre de 160 000 victimes par an pour les seules violences sexuelles commises sur mineur au sein du cercle familial, estimation probablement sous évaluée, ces violences étant par essence cachées et intimes.

Toutefois, et c’est le sens du rapport de notre collègue Marie Mercier, notre droit n’est pas dépourvu d’outils juridiques pour la protection des mineurs – Mme la ministre vient de le rappeler y compris dans des situations d’urgence, outils qui relèvent du juge des enfants, du juge aux affaires familiales ou du procureur de la République. Dans un premier temps, nous nous sommes donc demandé si le juge des enfants n’avait pas toutes les compétences requises pour protéger un enfant, sans avoir besoin de ce texte. le juge des enfants que nous avons entendu en audition nous a expliqué qu’il ne pouvait intervenir que lorsque les deux parents étaient défaillants et qu’il ne pouvait confier l’enfant à un parent protecteur. C’était donc bien au juge aux affaires familiales d’intervenir dans ce cas. Nous nous sommes donc tournés vers ces juges qui, eux, nous ont expliqué que l’assignation à bref délai et l’ordonnance de protection pouvaient déjà servir à cela et qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter une couche de procédure supplémentaire.

En effet, l’assignation impose au juge de statuer sur le fond dans l’urgence, ce qu’il ne peut pas toujours faire et ce qui conduit certaines juridictions surchargées à émettre un refus systématique.

Pour autant, cet outil est principalement destiné à la protection du conjoint victime, les enfants du couple n’étant alors concernés qu’à titre accessoire. Ainsi, dans le cas où les violences ne s’exerceraient que sur les enfants,

actuels, elle propose d’élargir le dispositif de l’ordonnance de protection aux cas vraisemblables de violences commises dans le cercle familial proche à l’encontre d’un enfant. L’ordonnance de protection deviendrait ainsi l’outil général de protection judiciaire d’urgence

La loi adoptée en mars dernier prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation.

Le juge aux affaires familiales doit pouvoir prononcer des mesures temporaires pour protéger l’enfant victime de violence, en statuant en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le principe de précaution a toujours guidé le magistrat appelé à délivrer une ordonnance de protection : les enfants devraient donc en bénéficier, tout autant que les adultes. La présomption d’innocence ne doit pas empêcher de prendre des mesures pour protéger en urgence l’intégrité physique et la santé mentale de l’enfant. Les enfants n’ont évidemment ni les ressources physiques, ni les ressources psychologiques, ni les ressources financières pour fuir un agresseur issu de leur propre cercle familial. Une mise en sécurité rapide, la plus précoce possible, est nécessaire, d’autant qu’il arrive très fréquemment que le parent mis en cause, tant qu’il n’est pas poursuivi en justice, ne soit pas éloigné de l’enfant.

Ne pas mettre en sûreté un enfant qui a dévoilé les violences qu’il a subies, c’est le dissuader de parler et le renvoyer au silence. Les enfants dénonçant les agressions dont ils sont victimes ne devraient jamais être laissés sans protection. Interdire au parent accusé d’entrer en contact avec l’enfant présumé victime est une avancée majeure quand on connaît les stratégies de manipulation des agresseurs. Ces derniers bénéficient souvent d’un niveau de protection et de crédibilité élevé au sein du cercle familial.

Dans la mesure où 88 % des violences incestueuses ne font pas l’objet d’une plainte, l’ordonnance de protection doit permettre de protéger l’enfant à partir d’un simple signalement, dès lors qu’il est à redouter que de nouvelles violences soient commises. Pour que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit pas qu’une formule creuse dans notre droit, nous devons nous doter d’outils plus ambitieux. La parole

à se livrer à des contorsions juridiques quelque peu risquées. Il est donc proposé que le juge aux affaires familiales puisse être saisi,

beaucoup trop souvent dans le cadre familial. Ainsi, l’instauration d’une ordonnance de sûreté spécifique aux enfants victimes de violences peut constituer une réponse juridique efficace, sur le modèle de l’ordonnance de protection en cas de violences conjugales. la société française, comme tant d’autres, s’est contentée de palliatifs, refusant de regarder en face la gravité des drames qui se jouent derrière les portes closes. Les chiffres, hélas ! parlent d’eux mêmes : 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. Chacune de ces vies est marquée à jamais ; ce n’est pas seulement un échec individuel, c’est aussi un échec collectif. La loi doit faire en sorte de protéger les membres les plus faibles de notre société, une catégorie à laquelle appartiennent nos enfants. La récurrence de ces drames et leur diffusion dans la société choquent la population et appellent une réponse judiciaire et pénale à la hauteur de l’émotion

Ce sont, chaque année, 160 000 jeunes victimes qui voient ainsi leur vie basculer. Parce que ce sont justement des enfants et que les violences subies se déroulent majoritairement dans le cadre familial, leur souffrance reste invisible ; il leur est en outre impossible Pour peu qu’ils soient frappés par un handicap, c’est encore pire : ils ont alors un risque 2,9 fois plus élevé d’être victimes de violences sexuelles. Lorsque leur handicap est lié à une déficience intellectuelle ou à une maladie mentale, le risque est 4,6

ci nous a convaincus, s’il en était encore besoin, de la nécessité d’agir sans faillir contre cette réalité terrifiante, non seulement en raison du coût social que ce fléau fait peser sur la société, mais surtout parce que le viol est un anéantissement de l’être et que l’impunité des violeurs d’enfants est absolument intolérable. Il nous a aussi rappelé combien il est nécessaire d’entendre la parole de l’enfant en toutes circonstances, selon l’adage « je te crois, je te protège », pour lui permettre de sortir de ce néant absolu. Trop souvent, malheureusement, l’accompagnement fait défaut, à tel point que le juge Durand parle d’un second anéantissement. L’absence de soutien social correspond selon lui à répondre « tu mens » à la malheureuse victime. Certes, de nombreuses initiatives ont vu le jour en matière de lutte contre les violences sexuelles sur les enfants. Je pense notamment au plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020 2022, qui a renforcé le 119 et qui a permis le contrôle systématique des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles exerçant une activité en contact avec des mineurs. Je pense bien évidemment à la création de la Ciivise ou à l’adoption, en 2021, de la loi Billon visant à protéger les mineurs des crimes et L’initiative de notre collègue Maryse Carrère s’inscrit dans cet esprit. La proposition de loi que nous examinons cet après midi entend créer un nouveau dispositif de protection judiciaire de l’enfant victime de violences. Toutefois, l’intérêt d’instituer une ordonnance de sûreté de l’enfant est apparu limité à notre commission des lois, d’une part, parce que le droit en vigueur répond déjà largement aux objectifs de ce texte, d’autre part, parce que la proposition de loi comporte moins de mesures de protection que celles dont dispose le juge aux affaires familiales lors de l’octroi d’une ordonnance de protection. En outre, contrairement à l’ordonnance de protection, aucune sanction pénale n’a été prévue en cas de violation des mesures prononcées par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de sûreté. La portée du texte s’en trouve, de ce fait, considérablement amoindrie. C’est la raison pour laquelle Maryse Carrère nous proposera un amendement de réécriture de l’article unique qui permettra d’atteindre le même objectif de protection de l’enfant victime de violences, mais dans le cadre d’une ordonnance de protection élargie de violences commises dans le cercle familial proche et nécessitant, par suite, une protection judiciaire d’urgence. Madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe souscrit pleinement à l’objectif qui sous tend cette proposition de loi. Nous saluons l’initiative prise par notre collègue pour ajuster son texte et enrichir le dispositif de l’ordonnance de protection, afin d’y inclure les violences sur les enfants, notamment sexuelles. C’est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de la proposition de loi ainsi amendée. Seuls comptent pour nous l’efficacité de la réponse,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi visant à instituer une ordonnance de sûreté spécifiquement dédiée aux enfants victimes de violences, lesquels méritent sans nul doute une attention particulière.

ce travail de fond met en lumière certaines faiblesses significatives du mécanisme envisagé. Tout d’abord, la pertinence même d’une ordonnance spécifique, intitulée ordonnance de sûreté, demeure incertaine. De nombreux dispositifs existent déjà, tant en matière de protection judiciaire de l’enfance que dans le cadre de l’autorité parentale. Plusieurs de ces dispositifs ont, du reste, fait l’objet de réformes récentes, notamment cette année au au travers de la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, qui a permis d’élargir les motifs de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la proposition de loi qui nous est soumise présente une redondance notable avec les mesures d’assistance éducative. En effet, les ordonnances de protection, ainsi que les autres prérogatives du juge aux affaires familiales, peuvent d’ores et déjà être activées pour protéger un enfant victime ou en danger.

leur réticence sur le fondement de considérations essentielles : ils regrettent l’absence de sanctions en cas de violation des mesures prononcées, un cadre juridique inadapté, ainsi qu’une potentielle atteinte à la lisibilité et à l’efficacité des dispositions en vigueur.

de l’enfance, au regard des évolutions importantes que celle ci a déjà connues ces derniers mois. Une évaluation de l’application des lois récemment votées permettrait, dans un premier temps, de mesurer leur impact réel et d’envisager, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Prendre le temps de cette évaluation est essentiel si nous voulons garantir des dispositifs durables, adaptés et pleinement fonctionnels. Mes chers collègues, notre volonté collective est de lutter contre les violences faites aux enfants. Cependant, ce qui est envisagé dans le cadre de cette proposition de loi ne garantit ni l’efficacité ni la pertinence du dispositif. C’est pourquoi nous nous en remettrons à l’avis de la commission. La parole

Je le dis et je le répète, la protection de l’enfance ne saurait être un concept abstrait. Elle ne doit pas être la variable d’ajustement de nos politiques sociales. Des dispositifs existent, qu’il s’agisse des ordonnances de protection, de l’autorité parentale adaptée ou encore des placements d’urgence.

permet au juge aux affaires familiales de prononcer en 24 heures des mesures de protection, comme l’interdiction de contact pour l’auteur présumé, la suspension du droit de visite et d’hébergement et des restrictions de déplacement.

et l’ordonnance de protection, moins lisibles et plus difficiles à mettre en œuvre pour les victimes comme pour les acteurs judiciaires. C’est pour cette raison que j’ai déposé un amendement de réécriture.

Ciivise nous le rappelle : l’urgence est non pas de voter de nouvelles lois, mais d’assurer l’application effective des textes existants. Ce que nous devons garantir, ce sont des moyens concrets pour que nos magistrats, nos éducateurs et tous les professionnels engagés dans la protection de l’enfance puissent agir.

un effort d’information et de prévention, car la loi et les juges qui l’appliquent ne peuvent pas tout. Parce que les enfants ne sont souvent pas capables de témoigner sur le moment des violences qu’ils subissent,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la protection des enfants victimes de violences est une priorité absolue pour notre société.

Ces dernières années, nous avons considérablement renforcé le cadre juridique de la protection des enfants. La loi du 18 mars 2024, dite loi Santiago, a ainsi élargi les motifs de suspension et de retrait de l’autorité parentale, permettant d’intervenir plus efficacement en cas de danger pour l’enfant. Ces réformes témoignent d’une volonté constante de mieux protéger les mineurs grâce à des outils éprouvés, comme l’ordonnance de protection ou les mesures d’assistance éducative prises par le juge des enfants. Ces dispositifs, bien qu’imparfaits, constituent aujourd’hui le socle de notre action.

Contrairement à l’ordonnance de protection, elle ne prévoyait aucune sanction en cas de non respect des mesures décidées par le juge, ce qui aurait pu limiter son effectivité.

des violences exercées par un parent, son conjoint ou son concubin. L’amendement de Mme Carrère vise à faire de l’ordonnance de protection un outil central de protection judiciaire d’urgence, pour répondre efficacement aux cas de danger manifeste. Pour garantir une mise en œuvre adaptée à la protection des enfants, plusieurs ajustements sont proposés. Premièrement, le dépôt d’une plainte pénale devient obligatoire, car un enfant ne peut agir seul en justice. Cette procédure permet de garantir que des démarches judiciaires soient engagées pour protéger la victime. le port d’un bracelet antirapprochement est écarté dans les cas impliquant des enfants, ce dispositif n’étant pas considéré comme adapté. Pour ces derniers, les situations d’urgence peuvent être traitées par d’autres moyens existants, comme la garde à vue d’un parent violent ou l’ordonnance de placement provisoire, délivrée par le procureur.

d’assurer une fluidité optimale entre les différentes autorités judiciaires impliquées, à commencer par les juges aux affaires familiales et les procureurs, et les autres acteurs de la protection de l’enfance. Le but ultime doit rester la sécurité de l’enfant, garantie par un système fiable, efficace et capable de répondre rapidement à toutes les situations de danger. La discussion générale

Hormis la demande d’assistance éducative, qui peut prendre la forme d’une requête, et non d’une plainte, émise par le mineur en danger, tous les dispositifs de protection judiciaire de l’enfance respectent ce principe. Il revient soit au parent protecteur, soit, en l’absence de ce dernier, au procureur de la République ou à un administrateur, de saisir, selon les cas de figure, le juge En matière pénale, les associations de défense des droits des enfants peuvent également porter plainte pour des faits de violences commis sur un enfant, conformément à l’article 2 3 du code de procédure pénale.

appel. Évidemment, cette incapacité à agir ne signifie pas pour autant que l’enfant victime de violences ne peut rien faire. Il peut, sans formalisme particulier, se signaler à la justice, notamment au parquet, et être entendu dans le cadre des procédures le concernant.

Quel que soit son lien de parenté avec l’enfant, l’agresseur est souvent protégé par la famille, qui veille à ce que le silence ne soit pas rompu. Une ordonnance de protection est donc nécessaire pour protéger l’enfant et lui permettre d’échapper à l’emprise de son agresseur,

Que ce soit à l’occasion d’une visite, d’une fête de famille ou de vacances, un agresseur a mille occasions d’exercer des violences sexuelles sans même habiter avec sa victime. Conditionner l’ordonnance de protection à la cohabitation serait donc très dangereux pour l’enfant. Au nom de la sécurité du mineur

Naminzo. Ce sous amendement vise à permettre la prolongation de l’ordonnance de protection au delà de douze mois, comme c’est le cas pour les femmes victimes de violences conjugales. La prolongation au delà de douze mois est, en tout état de cause, décidée par le juge aux affaires familiales. Celui ci devrait également pouvoir l’accorder aux enfants victimes de violences incestueuses. La protection et la sécurité d’un enfant ne peuvent être compromises par des délais de procédure trop longs.

Par ce sous amendement, nous proposons que les enfants puissent bénéficier de l’ordonnance provisoire de protection immédiate. Ce dispositif d’urgence, que nous avons adopté en juin dernier afin de protéger les femmes victimes de violences conjugales, est essentiel. Nous étions partis du constat suivant : chaque jour compte. Chaque jour où l’enfant risque de subir des violences est une perte de chance pour lui. La violence subie pendant l’enfance a un impact immédiat sur la scolarité et la capacité d’apprentissage des victimes. Le temps de l’enfance est un temps compté.

Aucune perte de temps ne saurait être admise, aucun risque de récidive ne peut être pris. Il est donc essentiel que les enfants puissent bénéficier de ce dispositif d’urgence.

En élargissant le champ de l’ordonnance de protection aux cas des violences familiales, et non plus aux seuls cas de violences au sein du couple, nous évitons la superposition des dispositifs de protection judiciaire. L’ordonnance de protection devient un dispositif général de protection des victimes présumées, qu’elles soient mineures ou majeures.

Je note, par ailleurs, que l’amendement apporte des adaptations au dispositif de l’ordonnance de protection pour tenir compte de la spécificité des violences commises à l’égard des seuls enfants. Je pense en particulier à l’obligation du dépôt de plainte, à l’impossibilité d’ordonner le port d’un bracelet antirapprochement, ou encore à l’irrecevabilité d’une demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate,

Concernant le sous amendement n° 14 et l’amendement n° 12 rectifié, qui n’est pas tout à fait identique à l’amendement n° 1 rectifié, le dépôt d’une plainte me semble un corollaire indispensable,

contre les seuls enfants. Cette procédure d’extrême urgence sans contradictoire me paraît inadaptée, dès lors qu’un parent protecteur est présent, condition nécessaire à l’octroi de l’ordonnance de protection. Sans cela, ce sont les ordonnances de placement qui sont pertinentes. Quel est l’avis

Ma seconde réserve vient du fait que le droit positif permet déjà au juge aux affaires familiales de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

de fait. C’est déjà le cas, puisqu’il revient d’abord aux parents de protéger leur enfant. Si l’intervention des parents, titulaires de l’autorité parentale, n’est pas suffisante, alors c’est au parquet ou au juge des enfants de prendre les décisions.

Ne parlons pas non plus de la compétence du juge des enfants, car, que je sache, nous ne proposons pas systématiquement que l’enfant soit placé. Le placement à domicile n’est en effet pas possible,

de l’inceste a permis d’établir des règles claires et strictes en matière de consentement. En deçà de l’âge de 15 ans, et de celui de 18 ans en cas d’inceste, toute relation sexuelle avec un adulte est désormais considérée comme un viol. Malgré cette avancée, les victimes sont encore confrontées à des parcours de protection et d’accompagnement fragmentés. Des dispositifs existent, et il est essentiel de renforcer leur accessibilité et leur efficacité. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 13 juin 2024, qui vise à améliorer la protection des victimes de violences intrafamiliales, mais dont le décret d’application demeure malheureusement en attente de publication. J’insiste sur l’urgence de le publier, pour ne pas retarder davantage la mise en œuvre de ces mesures. Il y a un an, la Ciivise a formulé quatre vingt appelant à des actions judiciaires plus adaptées, mais aussi à des mesures de prévention, de formation et d’accompagnement. Je tiens à cet égard à saluer le travail remarquable de son ancien coprésident, le juge Édouard Durand, et son investissement constant. Il incarnait une figure d’espoir pour les 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles. Je le rappelle, il y a une victime toutes les trois minutes ! Face à ces chiffres terrifiants, je salue l’initiative du groupe RDSE et de sa présidente, ainsi que les travaux de la rapporteure. si la proposition de loi que nous avons examinée aujourd’hui est évidemment intéressante, elle demeure insuffisante. Les initiatives s’accumulent et les textes se superposent nous devons veiller à leur cohérence. La méthode du pas à pas ne suffit plus. Le Gouvernement doit se saisir des recommandations de la Ciivise et travailler avec le Parlement pour bâtir un système de protection pleinement opérationnel contre les violences sexuelles. Personne ne

que, dans notre République, les malfrats bénéficient de droits auxquels n’ont pas accès les honnêtes citoyens ? Pour moi, la réponse à cette question est : non ! Tel est l’objet de la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous présenter, et qui vise à lutter principalement contre le blanchiment des espèces. En France, le code monétaire et financier précise les plafonds de paiements en espèces pour les transactions entre particuliers, entre professionnels, mais aussi entre particuliers et professionnels. Les textes limitent le paiement en liquide à 1 000 euros, énumérant des exceptions aux articles L. 112 6 à L. 112 8. Ainsi, le paiement en espèces entre particuliers n’a pas de plafond, mais il doit être régularisé par écrit au delà de 1 500 euros.

Selon la loi, ceux qui ne disposent pas de compte bancaire peuvent, en revanche, régler sans limitation de montant n’importe quel achat ou loyer en espèces. Les honnêtes gens peuvent à peine acheter un vélo d’occasion, alors que les voyous peuvent acquérir une berline de luxe ! Qui sont exactement ces 440 000 personnes concernées parce qu’elles n’ont pas de compte en banque ?

À mesure que le narcotrafic s’étend sur tout le territoire français, avec son lot de « narchomicides », il est aussi pourvoyeur de transactions records en espèces et, par la même occasion, de croissance de notre PIB.

sous couvert d’harmonisation de la réglementation européenne. L’argent n’a pas d’odeur – on le savait, et cela se confirme –, mais le narcotrafic est tentaculaire et frappe autant les villes que les territoires ruraux.

y pointent du doigt la nécessité de contrôler les flux d’argent liquide. Ce rapport décrit la multiplicité des méthodes de blanchiment des revenus du narcotrafic : réutilisation directe des fonds criminels ; réinjection des espèces dans le travail dissimulé

évitement du circuit bancaire… Autant de procédés facilitant l’extraction rapide des liquidités, devenues opaques, intraçables et insaisissables : 47 % des flux financiers produits par ces avoirs criminels sont constitués d’argent liquide, mais personne ne sait ce qu’il en advient. Avec cette proposition de loi, je m’attache à l’aspect monétaire du trafic. Les malfrats utilisent les espèces, par exemple, pour louer de grosses berlines, acheter des produits de luxe, installer des commerces, mais aussi pour corrompre. Aucune profession n’est épargnée, en particulier dans les ports et les aéroports où l’on corrompt certains agents. En avril 2023, le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale révélait d’ailleurs que plus de 90 % des billets de banque circulant aujourd’hui en France – y compris ceux que nous avons en poche

Mais alors, comment se fait il que des personnes dépourvues de ressources connues roulent encore au volant de grosses berlines ? Je vois un autre écueil financier, qui est le comble du cynisme. Lutter contre le paiement en espèces entraînerait immanquablement une baisse du PIB au vu des sommes concernées, ce qui augmenterait les ratios de la dette et des prélèvements obligatoires ! Mais, je le répète, l’argent n’a pas d’odeur… S’agirait il de la véritable raison de l’opposition que rencontre cette proposition de loi dans les sphères financières ? Je m’interroge

En effet, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent deux fléaux majeurs que notre appareil législatif doit impérativement combattre, en s’adaptant en permanence à l’évolution des risques et des pratiques frauduleuses. La crise que traverse actuellement notre pays en matière de narcotrafic, dont nous aurons l’occasion de débattre l’année prochaine, constitue l’un des aspects de cette problématique. Il est impératif que nous employions tous les moyens pour neutraliser les instruments de blanchiment de capitaux. Je rappelle, à cet égard, que les services répressifs ont procédé l’année dernière à plus de 24 000 saisies d’espèces pour un montant de près de 100 millions d’euros. C’est à ce titre C’est à ce titre que l’usage des espèces peut constituer un risque. En tant que moyen de paiement anonyme, facile d’utilisation et instantané, la monnaie fiduciaire peut, dans certaines circonstances, présenter un risque de blanchiment de capitaux. l’argent liquide constitue également un moyen de paiement auquel nos compatriotes demeurent largement attachés et qui n’est en aucun cas synonyme de blanchiment d’argent. Pour répondre au risque réel que représente la monnaie fiduciaire, le droit actuel prévoit déjà un encadrement strict des paiements en espèces. Cet encadrement, que je rappellerai, se doit d’être strictement proportionné dès lors qu’il entre en conflit avec le droit du paiement en espèces, lequel est l’expression directe du fait que les pièces et billets de banque ont cours légal dans la zone euro et qu’un commerçant ne saurait les refuser comme moyen de paiement sans motif légitime. Dans sa rédaction actuelle, le code monétaire et financier a prévu un seuil de droit commun de 1 000 euros pour les paiements en espèces effectués par les résidents. Au delà de cette somme, les résidents français ont l’obligation de recourir à un autre moyen de paiement. Pour les étrangers de passage en France qui, par construction, peuvent être amenés à transporter davantage d’argent liquide, un seuil aménagé à hauteur de 10 000 ou 15 000 euros est prévu dès lors que le paiement n’est pas effectué dans un cadre professionnel. Il faut relever ici que le plafond applicable en France, qui a été ramené de 3 000 à 1 000 euros en 2015, est l’un des plus robustes de la zone euro. En Belgique ou aux Pays Bas, ce seuil est trois fois plus élevé, tandis que dans plusieurs pays de la zone euro, parmi lesquels figurent l’Allemagne et la Finlande, aucun plafond n’est fixé pour les paiements en espèces.

Enfin, le code monétaire et financier prévoit deux exceptions générales, dont l’objet est de limiter la restriction au droit de payer en espèces pour les situations dans lesquelles le risque de blanchiment n’est pas caractérisé. pas caractérisé. Il s’agit, d’une part, des paiements entre particuliers pour des opérations non professionnelles et, d’autre part, des paiements des personnes non bancarisées, c’est à dire n’ayant pas de compte bancaire ou ne pouvant s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement. J’en viens aux mesures prévues dans la proposition de loi, qui sont fondées sur un objectif légitime de renforcement de la lutte contre la criminalité financière. Le texte prévoit d’abord de fixer un plafond spécifique pour le paiement des loyers. ensuite à supprimer le déplafonnement des paiements pour les opérations non professionnelles entre particuliers. Il vise enfin à supprimer le déplafonnement des paiements pour les personnes non bancarisées. Sur les deux premiers points, je relève que les loyers sont déjà soumis, en l’état actuel du droit, au plafond de droit commun de 1 000 euros. Quant aux paiements entre particuliers pour une opération non professionnelle, ils font partie des dépenses de la vie courante qu’il n’est pas souhaitable de réglementer dès lors qu’ils ne constituent pas une voie de blanchiment d’argent. Sur le troisième point, la commission a estimé après réflexion que la mesure proposée avait un caractère disproportionné. Je comprends l’intention de l’auteur de la proposition de loi, qui est d’empêcher tout contournement du droit en vigueur. des services chargés de la lutte contre la criminalité financière que j’ai entendus m’ont tous confirmé qu’ils n’avaient rencontré aucun cas documenté de contournement de la loi par un refus calculé d’ouvrir un compte bancaire. Peut être pourrez vous nous confirmer cette information, madame la secrétaire

Sur ce point, je tiens également à souligner l’existence d’une réglementation transversale antiblanchiment dont l’effectivité est assurée par Tracfin, notre cellule nationale de renseignement financier, est particulièrement efficace. L’obligation faite aux professionnels assujettis de réaliser un signalement à Tracfin en cas de soupçon de fraude est un instrument majeur qui permet, en l’état actuel du droit, de lutter contre les cas, envisagés par les auteurs de la proposition de loi, de paiements massifs en liquide, par exemple

Je remercie donc son auteur, Christian Bilhac, de permettre aujourd’hui cet échange de vues sur ce sujet important. En axant vos travaux sur les paiements en espèces, monsieur le sénateur, vous faites entrer la vie courante dans ce débat qui peut paraître de prime abord plutôt technique. Le Gouvernement partage, bien sûr, pleinement l’objectif de s’assurer que nos moyens de contrôle et d’encadrement soient, à tout moment, les plus efficaces possible. La criminalité financière évolue, et elle évolue rapidement. Face à ce constat, il est impératif que nous soyons réactifs si besoin, le cadre réglementaire. Le texte comporte trois évolutions principales, avec l’objectif que les paiements en espèces entre particuliers pour des opérations non professionnelles ne puissent pas constituer un canal de blanchiment des capitaux. prévoit de plafonner à 1 000 euros les paiements en espèces entre particuliers lorsque le débiteur est résident fiscal en France. Il s’agit d’une évolution majeure par rapport à la situation actuelle. Il existe en effet actuellement un plafond de 1 000 euros lorsque l’opération a lieu entre un particulier et un professionnel, mais il n’y a aucun plafond lorsque les personnes n’agissent pas pour des besoins professionnels.

Deuxièmement, le texte vise à supprimer la tolérance dont bénéficient aujourd’hui les personnes n’ayant pas de compte de dépôt. En effet, celles ci peuvent actuellement payer en espèces au delà du plafond de 1 000 euros prévu pour les titulaires d’un compte bancaire. Sans cette dérogation, lesdites personnes, souvent souvent fragiles – il est important de le rappeler –, seraient très pénalisées dans leur vie quotidienne. Troisièmement, la proposition de loi prévoit de mettre en place un parallélisme entre les règles applicables aux salaires et celles qui sont applicables au paiement du loyer entre particuliers un loyer de 1 500 euros ne pourrait plus être réglé en espèces entre particuliers. Ces différentes mesures ont le mérite d’ouvrir le débat, mais elles risquent, selon nous, de ne pas atteindre l’objectif de la proposition de loi.

L’absence de limite aux paiements en espèces entre particuliers est compensée par de multiples limites et contrôles à l’entrée de ces espèces dans le circuit économique. J’en citerai quelques unes. Il n’est par exemple pas possible en France de payer ses créances publiques en espèces au delà de 300 euros. Quant aux mouvements d’espèces aux frontières, ils sont surveillés, avec l’obligation pour les voyageurs de déclarer tout transport d’espèces supérieur à 10 000 euros.

euros. Enfin, au niveau européen, le règlement qui va entrer en vigueur en 2027 ne prévoit pas de plafond pour les opérations entre particuliers, particuliers, car la lutte, légitime, contre le blanchiment et le financement du terrorisme est d’abord une affaire de transactions entre professionnels. L’harmonisation des pratiques à l’échelle européenne est un excellent moyen pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce règlement introduira un plafond à 10 000 euros, alors qu’il n’en existe aucun aujourd’hui lorsqu’un professionnel est en jeu. Au niveau français, donc, des limites existent déjà. Elles sont en cours d’élaboration au niveau européen. Par ailleurs, ni la police judiciaire, ni Tracfin, ni les services du Trésor n’identifient de risques de blanchiment à la hauteur prévue dans cette proposition de loi. Le paiement des loyers entre particuliers ne semble pas représenter un outil de blanchiment. Dès lors, introduire un plafond à 1 500 euros n’est pas n’est pas un outil attendu et utile en la matière, alors que ce plafond représentera une gêne ou un obstacle pour les Français qui souhaitent régler en espèces en toute légalité. Ensuite, interdire tout paiement en espèces entre particuliers au delà de 1 000 euros ne peut être effectif que s’il est possible de contrôler ces transactions. c’est bien entendu impossible, et ce n’est même pas souhaitable, sauf à ce que l’administration soit particulièrement intrusive. il y a un risque réel, avec un tel plafond, que soient pénalisées les plateformes de revente en ligne ou de fourniture de services ponctuels entre particuliers, et avec eux une forme d’économie circulaire

Leur nombre est certes faible au regard des dizaines de millions de comptes bancaires ouverts en France, mais il n’est pas du tout négligeable. Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre droit encadre déjà le paiement en espèces, dans une perspective de lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le travail dissimulé.

L’argent liquide est un moyen de paiement crucial pour les personnes contraintes de recourir à un travail de subsistance, qui exercent des activités aux marges du salariat ou de l’activité indépendante. On estime que, en France, 3 millions de personnes vivent en situation d’exclusion financière.

aux personnes qui, faute de pouvoir payer de manière dématérialisée, n’auront plus accès au parc locatif. Ainsi, ce texte risque de marginaliser encore davantage les catégories de la population les plus fragiles économiquement.

L’argent liquide représente un coût que le secteur bancaire veut raboter, afin de faire des bénéfices en fermant des agences, pour substituer aux personnels des applications permettant un contrôle et une surveillance accrue des interactions avec les clients, le tout au profit des sociétés de paiement, qui pèsent désormais plus de 230 milliards d’euros. Alors que nos dépenses quotidiennes touchent à l’intime, se diriger vers le seul paiement dématérialisé provoquerait une véritable explosion

la société sans numéraire est l’une des formes les plus abouties du capitalisme de surveillance, car elle implique que chaque transaction passe par un complexe de banques, de sociétés de cartes, de fournisseurs de téléphonie et d’applications de paiement. accordons à ces sociétés financières un contrôle total sur le système monétaire, toutes nos interactions économiques seront enregistrées sur des bases de données privées, pour analyse. Enfin, il faut ajouter à ces risques qui concernent notre vie privée les points de défaillance de la dématérialisation. Alors que nos vulnérabilités se multiplient face au réchauffement climatique et qu’elles sont renforcées par l’absence de planification énergétique comme de souverain,

vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude en limitant les paiements en espèces. Elle tend notamment à réduire le seuil des transactions en espèces à 1 000 euros, à interdire le paiement des loyers en liquide et à supprimer les exemptions pour les personnes sans compte bancaire.

En revanche, elle affecterait durement certains de nos concitoyens et concitoyennes, en particulier les personnes les plus vulnérables. Le recours aux espèces reste aujourd’hui une réalité pour de nombreux ménages en difficulté, qui utilisent l’argent liquide non seulement comme moyen de paiement, mais aussi comme réserve de valeur. Supprimer les dérogations

compliquent l’accès aux services financiers, rendant ce droit souvent très théorique. Exiger de personnes précarisées qu’elles trouvent d’autres moyens de paiement que l’argent liquide pour les transactions supérieures à 1 000 euros, y compris pour le paiement des loyers, pourrait accentuer leurs difficultés et, dans certains cas, accélérer leur exclusion.

requis au delà de 1 500 euros. Imposer un tel plafond pourrait restreindre des habitudes de paiement courantes, comme lors de ventes de biens d’occasion ou de prêts informels. En limitant cette liberté, la loi risquerait de pénaliser des pratiques ordinaires qui, jusqu’ici, ne font pas l’objet de soupçons d’illégalité.

Au delà de ces considérations, la liberté des paiements en espèces relève de la philosophie politique. Est ce le rôle d’une société libérale que d’imposer un contrôle aussi renforcé des échanges monétaires entre acteurs économiques, nous rapprochant ainsi de la société de surveillance globale ? objectifs de la proposition de loi soient louables, ses mesures doivent être examinées avec prudence. La lutte contre la fraude et le blanchiment est essentielle, mais elle ne doit pas être menée au détriment des populations les plus fragiles. Pour toutes ces raisons,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre collègue Christian Bilhac, qui vise à limiter le paiement en espèces. Son but est de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et les activités criminelles connexes, telles que le trafic de stupéfiants ou la traite d’êtres humains. Ce texte modifie le code monétaire et financier en vue d’interdire l’utilisation des espèces pour le règlement des loyers au delà d’un seuil. Il prévoit aussi de supprimer les exceptions permettant des paiements supérieurs à 1 000 euros pour les transactions entre particuliers et pour les personnes non bancarisées. L’objectif affiché est de mieux contrôler l’usage de l’argent liquide, qui peut constituer un levier de fraude et de blanchiment. Nous y souscrivons tous, mais il est légitime de se demander si les mesures proposées sont vraiment efficaces et adaptées. Surtout, nous devons réfléchir à leurs impacts, notamment sur les populations les plus précaires. Pour commencer, rappelons que, selon la Banque de France, les espèces représentent encore 50 % des transactions aux points de vente en France,

en espèces est particulièrement visible chez les plus précaires, pour qui l’argent liquide est un outil indispensable de gestion de leur budget, surtout en période d’inflation.

Comme l’a souligné la Banque de France, de nombreuses personnes en situation de précarité éprouvent des difficultés à ouvrir un compte bancaire à cause de leur situation socio économique. En limitant le recours aux espèces, cette proposition de loi pourrait aggraver leur précarité et constituer pour elles une double peine. plus, la fixation d’un plafond pour les paiements en espèces des loyers soulève des questions. En effet, les services spécialisés dans la lutte contre la criminalité financière n’ont pas identifié de risques significatifs de blanchiment d’argent concernant ces transactions. de la suppression des dérogations pour les paiements en espèces entre particuliers. Là encore, les autorités compétentes n’ont pas relevé de risques notables en matière de blanchiment. Cela nous amène donc à nous demander si cette mesure sera vraiment efficace pour lutter contre les réseaux criminels. L’exposé des motifs cite l’exemple de la location de véhicules de luxe. Toutefois, ainsi que le rapporteur le souligne à juste titre, il serait plus pertinent de concentrer nos efforts sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, en imposant des obligations spécifiques aux professions concernées, plutôt que de prendre des mesures générales sur l’ensemble des paiements en espèces. Je souhaite également appeler l’attention sur un phénomène que nous constatons tous : le recul progressif de l’utilisation des espèces constitue un frein aux dons faits aux personnes sans abri, qui dépendent largement de ces gestes de solidarité pour survivre. En conclusion, bien que les objectifs affichés de cette proposition de loi soient tout à fait louables, on peut s’interroger sur l’efficacité de son dispositif. La suppression des dérogations pour les personnes non bancarisées ou pour les transactions transactions entre particuliers ne répond pas de manière adéquate aux problématiques du blanchiment et pourrait aggraver les difficultés des plus vulnérables. Dans ce contexte, bien que nous comprenions l’intention des auteurs de cette proposition de loi, nous estimons que les restrictions souhaitées ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre cette proposition de loi. La parole

La fraude fiscale nous empêche de financer nos politiques publiques. Outre les problématiques de santé publique qu’ils soulèvent, ces trafics ont donné lieu ces dernières années à de nombreux règlements de comptes entre bandes criminelles, provoquant autant de violences et d’insécurité dans nos villes et nos campagnes. Mes pensées aujourd’hui vont particulièrement aux populations marseillaises et grenobloises, qui ont connu cette année de nombreux

et la fraude fiscale. Lutte t on contre les trafics de drogue, contre la prostitution illégale, contre les braquages et l’évasion fiscale en interdisant à nos concitoyens d’utiliser leur argent pour les quelques usages où cela est encore permis ? Non, je ne le crois pas.

et de l’intérieur dans la lutte contre les fraudes. Restreindre la liberté de nos concitoyens dans l’usage de leur argent n’est pas une solution. Il s’agit là encore d’une ingérence supplémentaire de l’État dans le quotidien des Français. La libre utilisation de leur argent liquide est aussi un symbole de leur liberté. Certes, il ne s’agit pas d’être libertaire à outrance, mais l’utilisation des moyens de paiement liquides est déjà très largement encadrée. Par ailleurs, réguler l’utilisation de l’argent liquide ne permettra malheureusement pas de mettre fin

La société Chainalysis a estimé à cet égard que le volume des transactions illicites réalisées en cryptomonnaies, en premier lieu desquelles les fraudes et le blanchiment, a atteint 24,2 milliards de dollars en 2023

que d’utiliser leurs espèces pour vivre au quotidien. Les personnes âgées et ceux qui ne sont pas familiers du numérique – j’en fais partie ! – sont eux aussi les principaux utilisateurs de l’argent

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la lutte contre la criminalité financière constitue, à n’en point douter, une priorité unanimement partagée au sein de cet hémicycle.

La mobilisation collective autour de cet impératif a permis des avancées notables au cours des dernières années, parmi lesquelles figurent la réorganisation des services d’enquête de la douane française, le renforcement des moyens humains et financiers consacrés à la lutte contre la criminalité financière, et, plus récemment, la rénovation de la réglementation européenne le paquet de lutte contre le blanchiment des capitaux publié en juin 2024. La présente proposition de loi s’inscrit dans cet élan et mérite à ce titre d’être saluée. Son article unique vise à généraliser le plafond de paiement en espèces via la suppression de certaines dérogations. Une telle adaptation permettrait de s’assurer, selon son auteur, de l’absence de voies de contournement de la réglementation actuelle à des fins frauduleuses. Cette généralisation de la contrainte semble à première vue opportune. La question est légitime : pourquoi des pans entiers de la population seraient ils exonérés de ce plafond ? Aujourd’hui, les seuils d’autorisation de paiement en espèces font en effet l’objet d’aménagements pour tenir compte des particularités de certaines catégories de paiement. Parmi celles ci, trois dérogations sont en cause : le paiement des loyers, les transactions non professionnelles entre particuliers et les transactions effectuées par des personnes dites non bancarisées.

de certaines formes de criminalité financière. Toutefois, cette déduction mérite d’être confrontée à la réalité des faits. Les conclusions du rapporteur sont à ce titre pour le moins éclairantes aucun des experts auditionnés n’a permis de confirmer l’hypothèse d’une exploitation de ce régime dérogatoire comme vecteur de blanchiment. Les quelque 400 000 personnes non bancarisées en France sont en majorité dans une situation de grande précarité, qui ne leur permet pas de bénéficier de la politique de droit au compte bancaire mise en œuvre par la Banque de France. Dès lors, comment imaginer qu’ils puissent à loisir effectuer des transactions supérieures à 1 000 euros ? Si l’hypothèse de leur mise à contribution par les réseaux de blanchiment, en tant qu’intermédiaires, peut être envisagée, elle ne résiste pas à la réalité des faits.

Bien loin d’apporter une solution efficace à l’endiguement des pratiques de blanchiment, la présente proposition de loi augure donc d’une inutile complexification du régime dérogatoire actuel, mais aussi de restrictions des libertés manifestement disproportionnées.

vous séjournez à Amsterdam et vous tombez nez à guidon sur le vélo cargo de vos rêves ? Vous êtes de passage à Berlin et vous flashez sur une toile d’art contemporain ? Vous souhaitez faire l’acquisition d’un ordinateur sur un site de particulier à particulier ? Oui, mais vous vous souhaitez régler en espèces… Eh bien, prenez garde, car les plafonds autorisés pour ce type de transaction diffèrent d’un pays à un autre, d’un type de paiement à un autre. Sur la base d’un règlement de mai 2024 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux,

La proposition de loi de notre collègue Christian Bilhac vise justement un point précis : restreindre les possibilités de paiement en espèces au delà de 1 000 euros pour les particuliers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le code monétaire et financier définit en effet des plafonds pour les paiements en espèces suivant la nature de la transaction et la finalité professionnelle ou non de l’opération. Ainsi, le paiement des traitements et des salaires, d’une dette ou d’un prêt sur gage ne peut s’effectuer en espèces au delà d’un montant fixé par décret. Ce montant varie : pour les salaires, la limite est fixée à 1 500 euros ; pour une dette, elle est de 1 000 euros, sauf exception. ces dispositions ne s’appliquent pas aux transactions entre particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels, aux paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt.

La première vise à fixer un plafond spécifique pour le paiement des loyers, ces derniers étant actuellement soumis au plafond de droit commun de 1 000 euros. La deuxième tend à soumettre les paiements non professionnels entre particuliers au plafonnement de 1 000 euros prévus pour les résidents

du rapporteur : l’objectif serait plus efficacement atteint au moyen d’aménagements du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui assujettit certaines professions à des obligations spécifiques, plutôt que par des mesures générales concernant l’ensemble des paiements en espèces. de 400 000 personnes non bancarisées en France. Elles sont souvent dans une situation précaire qui ne leur permet pas de bénéficier de la procédure de droit au compte qui est ouverte par la Banque de France.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce n’est pas nouveau, le trafic organisé tue, la fraude fiscale fragilise notre pacte notre pacte sociétal, le travail dissimulé déstabilise notre économie et l’industrie du blanchiment d’argent alimente toute cette machine mortifère. Pour s’en convaincre, il suffit de considérer l’actualité inquiétante de ces derniers jours, liée aux conséquences tragiques du trafic de drogue : un jeune de 15 ans assassiné à Poitiers, une personne tuée à coups de couteau à Rennes ou encore un mort dans une fusillade à Valence. Quel est le point commun entre ces tragédies ? Leurs auteurs ont tous bénéficié directement ou indirectement du recours au paiement en espèces pour parvenir à leurs fins. Autrement dit, le paiement en espèces facilite le financement des activités illégales et constitue une véritable « malédiction du cash », pour reprendre les termes de certains économistes. En réponse, les mesures judiciaires et policières pour stopper les trafics en tout genre et la fraude fiscale sont indispensables. À cet égard, nous serons très attentifs au nouveau plan de lutte contre le narcotrafic présenté la semaine dernière par les ministres de la justice et de l’intérieur.

Une manne fiscale considérable échappe donc à l’État. Mes chers collègues, cela doit nous interpeller au moment où nous nous interrogeons sur l’avenir du financement du budget de l’État. Ne faudrait il pas mener aujourd’hui une évaluation de l’efficacité et du caractère complet de notre boîte à outils pour lutter contre ce phénomène ?

Dans une note publiée cet été, la Banque de France confirme qu’il existe un lien étroit entre la taille de l’économie souterraine et la demande de billets. Autrement dit, la régulation du paiement en espèces constitue un levier essentiel Dans cet esprit, la limitation des transactions en cash s’impose comme une réponse complémentaire et fondamentale à l’action judiciaire et policière menée par le Gouvernement, en particulier pour traiter le bas du spectre des activités illégales, qui reste pour l’instant sous les radars. En ce sens, la proposition de loi, présentée par notre collègue Christian Bilhac au nom du groupe du RDSE, apporte quelques solutions. En s’attaquant au financement des activités illégales, elle participe à la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif d’intérêt général suffisant

Le présent texte, proposé par Christian Bilhac, répond à une préoccupation qui nous est commune : le renforcement de l’efficacité de la lutte contre la criminalité financière. Cependant, si nous souscrivons à la volonté de lutter contre le blanchiment, l’article unique de cette proposition de loi ne constitue pas la voie adéquate pour atteindre cet objectif. Nous faisons nôtres les griefs exprimés par notre collègue rapporteur pour rejeter le texte. Ces trois mesures de restriction du droit au paiement en espèces risqueraient de complexifier le régime actuel et d’entraver certaines libertés individuelles, sans garantir de bénéfice réel en matière de lutte contre la criminalité financière. Premièrement, en ce qui concerne l’introduction d’un plafond spécifique pour le paiement des loyers, les services de la direction générale du Trésor n’ont pas identifié de risque significatif de blanchiment relatif au versement des loyers. De la même manière, le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme estime, lui aussi, que la menace de blanchiment liée à la location immobilière est faible au regard du cadre existant. Dès lors, introduire un nouveau plafond pour cette catégorie de transactions compliquerait le régime en vigueur, sans aucune certitude de renforcer la lutte contre la fraude. La seconde mesure, qui consiste à étendre le plafonnement de 1 000 euros au delà duquel le paiement en espèces est interdit aux transactions non professionnelles entre particuliers, apparaît quant à elle disproportionnée. Outre que, encore une fois, aucun risque particulier de blanchiment n’est lié à ce type de transaction, le plafond applicable constitue déjà l’un des seuils les plus stricts de la zone euro. Or le paiement en espèces reste le moyen privilégié pour les opérations entre particuliers. En restreignant cette liberté, nous risquerions d’entraver des transactions légitimes du quotidien, alors même que nous serions dans l’incapacité de vérifier l’effectivité de la mesure, puisque ces transactions ne font pas l’objet d’un contrôle systématique de l’administration. Enfin, la troisième et dernière mesure, qui consiste à soumettre les personnes non bancarisées au plafond de 1 000 euros, soulève un enjeu social important. 400 000 personnes ne disposent ni d’un compte bancaire ni d’un chéquier en France. De plus, ces citoyens sont souvent confrontés à la précarité, ce qui les écarte de la procédure de droit au compte mise en œuvre par la Banque de France. Dès lors, leur interdire les paiements de plus de 1 000 euros en espèces, alors même qu’ils n’ont pas de moyen de paiement de substitution, laisse poindre un risque important d’accroissement de leur précarité. En ce sens, supprimer le régime dérogatoire dont bénéficient les personnes non bancarisées nous semble disproportionné, d’autant que, je tiens à le rappeler, rien ne garantit qu’une telle mesure permettrait de renforcer la lutte contre la criminalité financière, dans la mesure où aucune corrélation entre les

Il nous faut continuer à combattre le blanchiment des capitaux issus de trafics illicites et, plus encore, veiller à ce que la réglementation actuelle ne soit pas contournée. Néanmoins, l’article unique de la présente proposition de loi ne permet pas d’atteindre les effets attendus par l’auteur du texte. Ainsi, nous rejoignons les craintes de notre collègue rapporteur quant à la mise en place d’un durcissement disproportionné de l’encadrement actuel du droit au paiement en espèces. En effet, nous ne saurions ignorer les indications des services du Trésor, qui n’établissent pas de lien entre, d’un côté, les transactions non professionnelles entre particuliers, le versement des loyers et les personnes non bancarisées et, de l’autre, la criminalité financière. Nous bénéficions d’ores et déjà d’un encadrement strict visant à lutter contre le blanchiment. Complexifier le cadre en vigueur, sans aucune garantie de tenir les résultats escomptés, nous semble contre productif. Cela nuirait à la clarté du dispositif, entraverait certaines libertés individuelles et risquerait de fragiliser les personnes non bancarisées. Pour l’ensemble de ces raisons, les sénateurs du groupe Union Centriste suivront la position

1 rectifié. Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi. Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi. Y a t il des demandes d’explication de vote ?…